Pour ces trois projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord instituant la Fondation internationale UE-ALC

armées est favorable à l'adoption de ce texte. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille

après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

de loi présenté permet la ratification de l'ordonnance 2017-1252 qui transposait la directive « DSP 2 » de 2015. La directive européenne n° 2015/2366, dite « services de paiement 2 », met à jour et complète le dispositif européen d'encadrement des services de paiement, en vue d'encourager cette activité dans le marché intérieur de l'Union européenne. Cette directive constitue ainsi une mise à jour de la directive du 13 novembre 2007 relative aux services de paiement, dite « DSP qui avait introduit un premier cadre d'activité en complétant la typologie des acteurs bancaires. Cette directive a notamment créé le statut d'établissements de paiement, complété en 2009 par le statut d'établissements de monnaie électronique. La reconnaissance d'un statut spécifique a permis le développement de ces services très usuels aujourd'hui grâce aux paiements en ligne. Ces acteurs bénéficient notamment d'un régime simplifié par rapport aux établissements de crédit. Quelles ont été les avancées permises par la directive DSP 2, dont nous achevons la ratification par ce projet de loi de ratification présenté aujourd'hui devant vous ? Premièrement, la directive complète le cadre juridique applicable aux prestataires de services de paiement supervision des prestataires de services de paiement, droits et obligations des parties à un service de paiement. Deuxièmement, elle élève les standards de sécurité des transactions, en particulier en généralisant le principe d'une authentification forte pour les transactions en ligne. Troisièmement, elle apporte une reconnaissance juridique à deux nouvelles catégories d'acteurs : les agrégateurs de comptes, qui offrent un accès pédagogique à l'information financière individuelle tant pour les entreprises que pour les particuliers ; les initiateurs de paiement, dont l'activité d'intermédiaire doit permettre de fluidifier la réalisation des virements. La traduction dans notre droit de cette directive constitue une opportunité pour la place financière française et s'inscrit pleinement dans les objectifs poursuivis par le Gouvernement favoriser l'innovation, renforcer la concurrence pour dynamiser la croissance, et améliorer les services rendus aux consommateurs et aux entreprises, tout en assurant un niveau de sécurité maximal des paiements. La France a toujours été à la pointe de l'innovation en matière de paiements- nous avons ainsi été pionniers dans le paiement par carte à puce. Elle doit le demeurer, et continuer de l'afficher. C'est l'ambition que nous nous sommes donnée au travers de cette transposition. Aussi le Gouvernement a-t-il souhaité transposer avec plusieurs mois d'avance cette directive, afin de permettre à l'ensemble des acteurs de la place de s'approprier ces nouvelles dispositions, d'asseoir la confiance du marché et d'attirer les innovateurs. européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur a ainsi été adoptée le 9 août 2017, avec près de six mois d'avance par rapport à sa date d'entrée en vigueur, faisant de la France l'un des premiers pays à transposer la directive, et le premier à avoir officiellement agréé un agrégateur de compte et initiateur de paiement. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Le projet de loi qui vous est soumis vise à procéder à la ratification de cette ordonnance par le Parlement. Le Gouvernement souhaite au travers de ce texte compléter le dispositif défini dans l'ordonnance sur deux principaux points : l'accompagnement du nouveau service de remise d'espèces lors du passage en caisse, dit « », et l'accélération

lors d'un achat, plus connu sous l'appellation « ». Ce service existe chez la plupart de nos voisins, par exemple en Allemagne, en Espagne, en Belgique et au Royaume-Uni. La directive « services de paiement 2 » indique que ce service peut, en théorie, être fourni sans être soumis aux règles prévalant pour les services de paiement. Elle laisse de fait très largement aux États le soin d'en définir les modalités pratiques d'exercice. Ce service présente de nombreux avantages sur lesquels je souhaite attirer votre attention. C'est un net progrès pour favoriser l'accès aux services financiers de base pour tous les Français, qui permettra de répondre à l'isolement des territoires les plus reculés, dont les relais d'accès aux espèces sont souvent trop limités ou éloignés. C'est un sujet sur lequel, je le sais, les élus locaux sont très mobilisés. C'est une opportunité de services nouveaux pour les consommateurs et pour les commerçants : ce service permettra d'attirer davantage de clientèle, par l'ouverture d'un service additionnel. Il offrira un moyen de gérer plus efficacement les encours en caisse pour les commerçants. Les associations de commerçants écoutées sur ce sujet ont souligné leur intérêt pour l'apparition d'un tel service. Le dispositif que nous proposons dans ce projet de loi permettra ainsi d'offrir un cadre lisible et stable pour les commerçants, afin d'encourager cette pratique, mais également d'assurer la qualité de la circulation de la monnaie fiduciaire sur l'ensemble du territoire et de prévenir les risques de blanchiment et de prévenir les risques de blanchiment en précisant ses modalités, par la fixation de seuils de retrait par voie réglementaire. En deuxième lieu, le Gouvernement

La directive DSP 2 prévoit que l'essentiel de ses dispositions entre en vigueur au 13 janvier 2018. La directive renvoie toutefois à une norme technique réglementaire, ou NTR, de l'Autorité bancaire européenne, l'ABE, un pan essentiel du dispositif, relatif aux modalités informatiques d'accès aux comptes de paiement par les nouveaux acteurs. Concrètement, cette norme technique détaille le fonctionnement des interfaces de communication sécurisées, appelées « API », par lesquelles ces acteurs pourront accéder, en pleine sécurité, aux données individuelles de comptes bancaires. Mais cette norme, qui a été publiée tout récemment, n'entrera en vigueur que 18 mois plus tard, soit en septembre 2019. Il nous semble que cette période transitoire peut engendrer des risques en termes de cybersécurité pour l'ensemble des acteurs, car elle conduit à pérenniser pendant cette durée la pratique actuelle dite du « », qui consiste, en récupérant les identifiants et mots de passe de l'usager, à accéder pour lui à son compte bancaire en ligne.

Il est donc proposé d'anticiper son entrée en vigueur, afin que, pour les banques prêtes en avance, l'API puisse être testée et rendue obligatoire, et ce dès la fin de 2018, si elle satisfait aux exigences de performance et de qualité définies par la norme technique et qu'elles assurent que les nouveaux acteurs tiers pourront continuer d'exercer leur pourront continuer d'exercer leur activité. Cette disposition a pour objectif de garantir la protection des utilisateurs de ce type de service. Enfin, et pour conclure, nous savons que la transposition de cette directive a suscité des questions sur les modalités d'exercice des nouveaux acteurs tiers, notamment lorsque ceux-ci accèdent aux données de comptes d'épargne. d'épargne. La directive DSP 2 se limite à encadrer l'accès, par les agrégateurs de comptes et initiateurs de paiement, aux comptes de paiement et ne traite pas de l'accès aux autres comptes- épargne, crédit, ou autres. Les négociateurs européens s'en sont tenus au champ qui avait été identifié par la directive, ce que l'on peut comprendre. Mais l'accès aux données sensibles des comptes tels que les comptes d'épargne ou les comptes titres mérite un cadre aussi sécurisé que celui qui est prévu pour l'accès aux données de comptes de paiement. Le nouvel article 1 introduit par le rapporteur et adopté par la commission des finances met le doigt sur cette difficulté. Le Gouvernement partage la volonté de soutenir les acteurs innovants tout en maîtrisant les risques attachés à leur activité pour ce qui dépasse le champ de la directive DSP 2. Toutefois, il nous semble que la réponse à cette question passe en premier lieu par une modification des textes européens. Le Gouvernement s'est engagé à lutter contre toutes les surtranspositions du droit européen à l'échelle nationale, notamment pour ce qui concerne le droit financier. La raison en est simple : alors que nous faisons des efforts importants pour renforcer l'attractivité de notre place financière en vue d'attirer davantage d'acteurs et d'institutions en France, notamment dans le secteur porteur des paiements, il serait peu compréhensible que nous imposions aux acteurs qui se développent chez nous des règles supplémentaires qui n'existent pas ailleurs. Or l'obligation de disposer d'une assurance de responsabilité civile professionnelle ou d'une assurance comparable associée à une obligation d'enregistrement engendre des formalités dont l'impact doit être soigneusement évalué, dans un contexte très concurrentiel au niveau européen. Ainsi, tout en rejoignant la préoccupation du rapporteur, il nous semble qu'un travail complémentaire est indispensable pour calibrer au mieux les modalités d'encadrement de l'accès aux comptes d'épargne, et sur cette base, pour engager dans les meilleurs délais une modification du droit européen. Nous devrons en effet réfléchir à une intervention au niveau national, sur la base d'une étude d'impact plus documentée que celle dont nous disposons aujourd'hui. À cet effet, nous engagerons une mission de réflexion pour formuler des propositions adéquates à porter auprès de nos partenaires européens et de la Commission européenne.

En effet, cette directive fait suite à une première initiative européenne qui, avec la directive « DSP 1 » du 13 novembre 2007, avait mis fin au « monopole » des banques sur la fourniture de services de paiement.

le Compte-Nickel, qui permettent d'offrir de nouveaux services à des populations qui étaient parfois éloignées des services bancaires traditionnels. Cette seconde directive, « DSP 2 », vise à prendre en compte les nombreuses évolutions survenues depuis 2007. Pour ne donner qu'un chiffre, 40

Dans ce contexte, la directive de 2015 encadre l'activité de ces nouveaux acteurs et améliore le fonctionnement du marché intérieur des paiements. À cet effet, elle poursuit quatre objectifs principaux reconnaître ces nouveaux acteurs et réglementer leurs relations avec les gestionnaires de compte et les utilisateurs ; renforcer les exigences de sécurité pour l'ensemble des paiements électroniques ; lutter contre le risque d'arbitrage réglementaire ; garantir un meilleur niveau de protection aux consommateurs dans leurs relations avec les prestataires de services de paiement. L'ordonnance prévoit une transposition globalement fidèle de la directive et fait bon usage des marges de manoeuvre laissées aux États membres. Sa ratification ne pose donc pas de difficulté.

La commission des finances est également favorable aux deux dispositions introduites par l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement. Il est en effet utile que le pouvoir réglementaire puisse fixer les modalités transitoires de communication sécurisée applicables en France jusqu'à l'entrée en vigueur des exigences de sécurités établies au niveau européen, afin d'accélérer la sécurisation des connexions entre prestataires et et gestionnaires de comptes. La commission des finances a toutefois précisé que les mesures réglementaires devraient respecter les normes techniques déjà prévues par l'acte délégué de la Commission européenne.

1 A. En effet, la directive « DSP 2 » fixe des règles strictes pour les agrégateurs de comptes et les initiateurs de paiement, en leur imposant à la fois l'obtention d'un agrément agrément ou de s'enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, et de communiquer avec le gestionnaire de compte par le biais d'un canal de communication sécurisé et standardisé.

la possibilité pour l'utilisateur d'obtenir un remboursement auprès du prestataire tiers en cas de fraude. La responsabilité des prestataires pourrait être engagée, ces derniers devant dès lors souscrire une assurance complémentaire

le 21 février dernier la conférence des présidents a demandé à la commission des affaires européennes d'exercer, à titre expérimental, une veille sur l'intégration des normes européennes en droit interne afin, notamment, d'informer le Sénat sur d'éventuelles surtranspositions. C'est donc avec cette préoccupation que la commission a examiné, sur le rapport de notre collègue Jean-François Rapin, qui est malheureusement retenu dans son département, le projet de loi ratifiant l'ordonnance de transposition de la directive sur les services de paiement. La deuxième directive sur les services de paiement, on le sait, entend favoriser l'innovation, la concurrence, l'efficience et la sécurité des services de paiement fournis au sein de l'Union européenne, afin d'élargir et d'améliorer les choix des consommateurs. Elle révise à cet effet les conditions d'agrément et d'exercice de ces services. Elle renforce les exigences de sécurité et de protection des données en imposant des normes techniques rigoureuses, comme l'« authentification forte » des clients, à compter de septembre 2019. Elle améliore les droits des utilisateurs de ces services. La commission des affaires européennes a formulé dans son rapport plusieurs observations sur la transposition à laquelle a procédé l'ordonnance. Tout d'abord, elle a constaté que, de manière générale, cette transposition était rigoureuse. Ensuite, elle a relevé que l'ordonnance avait retenu quelques-unes des facultés ouvertes aux États membres, par exemple l'allégement des conditions d'agrément et des exigences prudentielles auxquelles sont soumis les petits établissements de paiement, dont la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement est inférieure à 3 millions d'euros. Elle a également constaté que l'ordonnance faisait usage de la faculté ouverte par la directive d'imposer la désignation d'un point de contact central à tous les établissements de paiement agréés dans un autre État membre qui ont recours en France à des agents en libre établissement ou à des succursales. Ces points de contact faciliteront ainsi la supervision des activités transfrontalières. La directive encadre deux services de paiement connexes dits « tiers le service d'initiation de paiement et le service d'information sur les comptes, qui fournit au client une vue agrégée d'ensemble sur ses comptes de paiement et soldes disponibles. Elle soumet ces services à des conditions allégées d'enregistrement et de radiation et leur fait obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle ou une garantie comparable. Enfin, elle prévoit de leur ouvrir un accès sécurisé aux données utiles. Concernant l'agrégation des comptes, la commission des affaires européennes a observé que la directive ne couvre pas l'information sur des comptes autres que les comptes de paiement, en particulier les comptes d'épargne. Cela s'explique par le fait qu'elle ne concerne que le marché intérieur des paiements et les services de paiement. Or les comptes d'épargne constituent la part la plus importante- à hauteur de 80 %, comme l'a rappelé le rapporteur général -de la situation financière des personnes physiques. Dès lors, afin de pouvoir également agréger les soldes de ces comptes, les qui dispensent ce service utilisent les données de connexion que leur transmettent les titulaires pour collecter les données par voie de, c'est-à-dire de capture d'écran. Les risques associés à une telle pratique et l'absence de responsabilité des agrégateurs de ces comptes ont conduit la commission des affaires européennes et la commission des finances à s'interroger sur l'opportunité d'un encadrement de cette activité, et donc d'une extension de certaines dispositions de la directive à l'agrégation des comptes d'épargne. La commission des finances propose de procéder immédiatement à un encadrement minimal. Au-delà, la commission des affaires européennes estime que la France devrait porter sans tarder cette question au niveau européen, en concertation avec les teneurs de ces comptes, en particulier pour déterminer les exigences de sécurité et répartir la charge du financement de l'interfaçage. Cet exemple montre, si besoin est, que toute surtransposition n'est pas condamnable, mais doit être dûment justifiée.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, notre débat de ce jour est certes nécessaire, même s'il semble bien éloigné des préoccupations du jour, eu égard à la réalité d'un mouvement social multiforme mettant de plus en plus en question la logique gouvernementale à l'oeuvre depuis dix mois. Il s'agit d'assurer la transposition, dans le droit national, de directives européennes relatives aux services de paiement. Reconnaissons d'emblée à la commission des finances, à ses administrateurs et au rapport finalement produit, d'avoir créé de bonnes conditions de cette transposition, illustrées par les amendements déposés sur le texte transmis par l'Assemblée nationale. amendements s'avèrent, au-delà des dispositifs techniques nécessaires, utiles et n'appellent donc pas d'observations. Le sujet qui nous intéresse appelle tout de même quelques remarques, car nous sommes dans un univers bien précis : celui des secteurs financiers et de la banque en particulier. La directive pourrait en effet être limitée, dans la pratique, à une forme de facilitation du commerce en ligne, qui prévoit évidemment des formes de paiement dites « sécurisées » de plus en plus performantes, ou à la possibilité, en même temps qu'un plein d'essence, de pouvoir remplir son porte-monnaie de quelques espèces supplémentaires Je dois avouer que, sachant qu'il existe des logiciels de caisse quelque peu incertains, cette possibilité de retrait d'argent liquide en dehors des guichets bancaires et des distributeurs automatiques en fonctionnement laisse quand même certaines questions de sécurité en suspens. Revenons maintenant à l'essentiel, à savoir que le secteur bancaire a fait l'objet, dans la dernière période, de pressions fortes et que les évolutions s'y annoncent fondamentales. Prenons les données du problème. La Société générale a annoncé pour 2017 un bénéfice en baisse, mais s'établissant tout de même à 2,81 milliards d'euros. Le Crédit agricole, pour 2017, présente un bénéfice en légère hausse de 3,65 milliards d'euros, ce qui montre que la médiocrité du revenu moyen agricole ne semble pas perdue pour tout le monde Le groupe Banque nationale de Paris-Paribas, pour sa part, présente un résultat de 7,8 milliards d'euros, en progression d'environ 6,7 % par rapport à 2016. Le premier groupe bancaire de notre pays, considéré comme hautement systémique, présentait- il faut le dire -un résultat net bancaire de 43,4 milliards d'euros pour l'exercice 2016, somme qui semble prouver que la dette publique n'est pas perdue pour tout le monde Pour faire bonne mesure, la banque va distribuer un peu plus de 3,6 milliards d'euros en dividende à ses actionnaires. Dans le même temps, comme dirait l'autre, au-delà de ces situations financières qui montrent la bonne santé générale du secteur bancaire français, l'ensemble des réseaux est engagé dans un processus de réduction des des implantations et des effectifs employés. Ainsi, la Société générale entend réduire de 300 le nombre de ses agences sur le territoire, la réduction des implantations allant de pair avec celle des emplois correspondants. De même, le développement de la banque en ligne, évidemment moins mobilisateur de moyens, est privilégié, d'autant que l'opérateur historique des télécommunications s'est lancé dans l'aventure à son tour. Comme d'habitude, les banques en ligne ne sont jamais très éloignées des têtes de groupe bancaire, puisque B for bank n'est qu'un élément du groupe Crédit agricole, Hello bank, du groupe BNP-Paribas, que Boursorama est rattaché à la Société générale. Tout se passe donc comme si le produit net bancaire trouvait désormais son origine dans la dématérialisation des opérations, la réduction des réseaux « en dur » et des effectifs allant de pair avec ces réseaux. Ajoutons-y la facturation sans doute excessive de nombre de frais bancaires, ne serait-ce que ceux qui sont liés à la mise à disposition d'une carte de paiement sécurisée, et une intense campagne permanente en tant que « groupe de pression pour dégager les marges de manoeuvre indispensables à la poursuite de la rentabilité. Nous en avons d'ailleurs eu l'illustration récente puisque, après plusieurs années de travail sur l'assurance emprunteur pour mettre un terme aux ventes liées de contrats de prêts et de contrats d'assurance, nous avons vu réapparaître dans le texte sur la « société de confiance » la problématique du taux effectif global et celle du taux annuel effectif global. Sans doute un pur hasard, puisque, dans certains cas bien connus, la déchéance des intérêts a été acquise par des emprunteurs confrontés à l'absence d'indication de ces taux ... Je dois dire que le fait que les préoccupations bancaires aient ému le Gouvernement nous a quelque peu interpellés, surtout dans un texte destiné à rendre plus franches et plus loyales les relations entre administration et administrés. Je ne peux cependant terminer cette intervention sans revenir sur ce qui constitue, selon nous, la question principale de l'avenir de notre secteur bancaire et financier, en tout cas du point de vue du public. Que les banques soient amenées à jouer un autre rôle dans l'économie en finançant davantage qu'elles ne le font aujourd'hui les entreprises qui entreprennent, et pas uniquement celles qui montent de coûteux raids de prise de contrôle sur la concurrence, est bien entendu au coeur du débat. Mais il reste et demeure un sujet clef celui de l'accessibilité bancaire. Il est grand temps, mes chers collègues, que cette question trouve une solution plus honorable que l'actuelle législation, qui ne règle qu'une partie des questions. Le code monétaire et financier a sans doute besoin d'une évolution pour rendre effectif le droit au compte qui est, tout de même, essentiel pour éviter des signes d'exclusion sociale. que la commission des finances se penche quelque peu sur la question. C'est en tout cas l'intention de mon groupe. Pour le reste, nous n'avons pas d'opposition quelconque à l'adoption de ce projet de loi, somme toute assez technique. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les jours se suivent et ne se ressemblent pas puisque, hier, nous avons passé une grande partie de la journée à débattre des moyens de protéger nos données personnelles alors qu'aujourd'hui nous les ouvrons à grands bras pour ce qui concerne les services financiers.

je vous présenterai une intervention qui pourrait s'intituler « La directive marché intérieur pour les nuls ». Je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne, car le vocabulaire est assez technique et la pratique l'est tout autant. Finalement, si c'est assez simple, quand on y regarde de plus près, ça ne l'est pas tant

en ligne, en général par carte bancaire. Le PSP s'appuie sur des banques acquéreurs qui garantissent l'accès au réseau de paiement. D'après le code monétaire et financier, un prestataire de services de paiement est un établissement de crédit ou un établissement spécialisé dans les paiements, ce qui est une bonne chose, car à ce statut sont attachées des garanties

Les services d'initiation de paiement permettent au consommateur de demander à un intermédiaire de présenter et d'exécuter des opérations de paiements en leur nom auprès de leur banque. Voilà encore un intervenant

tout à fait heureux que la commission des finances ait adopté un amendement de protection et d'assurance. Mais, en réalité, avec un paiement unique, la durée de conservation des données court jusqu'à la réception du bien ou l'exécution de la prestation de service, augmentée du délai de rétractation prévu pour les ventes de biens ou de fourniture de prestations de services à distance.

Les données ainsi conservées à des fins de preuve peuvent être conservées en archive intermédiaire et n'être utilisées qu'en cas de contestation. Comment vérifier que nos données personnelles sont bien effacées de tous ces registres ?

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi dont nous avons à connaître aujourd'hui, qui ratifie l'ordonnance du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement dans le marché intérieur, est une étape importante de la construction d'un marché intérieur plus efficace et plus en phase avec la réalité et les perspectives de ce secteur d'activité. Car si le marché intérieur est une réalité depuis vingt-cinq ans, sans régulation des nouveaux acteurs et des nouvelles pratiques, son existence ne serait qu'illusoire. Cette directive, et le projet de loi qui en assure la transposition, cherche à concilier deux impératifs un niveau de sécurisation des données et des transactions conformes au plus haut standard, et l'ouverture de ce marché aux opérateurs de et à des modes de paiement alternatif. Applicable au 13 janvier 2018 pour une partie de ses dispositions et en août 2019 en ce qui concerne les dispositions techniques qui seront prises par décret, cette directive prévoit un certain nombre de modifications du droit qu'il est possible de synthétiser ainsi. Tout d'abord, l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur des paiements modifie la relation classique qu'entretenait la banque avec ses clients. Aujourd'hui, le développement des agrégateurs d'informations ou des initiateurs de paiement a conduit l'Europe à créer un encadrement distinct de celui qui est applicable aux banques. Ces initiateurs de paiement qui servent d'interface entre le client et l'entreprise en supprimant les moyens de paiement classiques que constituent la carte de paiement et le chéquier sont déjà très présents outre-Rhin. Quant aux agrégateurs d'information, à l'heure du, ils synthétisent l'ensemble des informations bancaires sur une interface indépendante des interfaces proposées par les banques. Le régime juridique de ces deux nouveaux types d'opérateurs se singularise par deux aspects : un régime d'enregistrement simplifié et une absence de contraintes en matière de capital minimal, cette dernière règle s'expliquant au regard de l'absence de détention de capitaux appartenant aux clients par ces organismes. Par ailleurs, face aux flux transfrontaliers de données bancaires, il est apparu important de renforcer la sécurité des données des consommateurs. En effet, cette directive cherche à limiter les risques d'asymétrie réglementaire, en empêchant du dumping technologique qui favoriserait les entreprises domiciliées dans des États moins-disants en termes de sécurité. Ainsi, elle rend obligatoire l'authentification réputée forte, c'est-à-dire l'authentification à deux facteurs, ou avec un mot de passe à usage unique. De plus, elle permet le développement de la technologie dite « API », qui permettra de davantage sécuriser les échanges d'informations entre les clients des banques et les nouveaux acteurs.

Il s'agit alors de « rendre la monnaie » lors d'un paiement par carte bancaire, les chèques étant exclus de cette procédure. Si ce type de pratique peut sembler étrange en France, pays qui a inventé la carte bancaire, elle constitue un mode alternatif de récupération de monnaie pour le consommateur sans passer par un distributeur. Là encore, un décret précisera ce dispositif et fixera un montant minimal de paiement ainsi qu'un montant maximal d'espèces pouvant être récupérées. Ce montant maximal ne peut être, dans notre esprit, qu'extrêmement limité.

les banques, elles, dépositaires des fonds des clients, souhaitent d'abord renforcer la sécurité, peut-être parfois au détriment de la rapidité d'accès. La position des banques s'explique puisque, en dernière analyse, il leur appartiendra de rembourser leurs clients, à charge pour elles de se retourner ensuite vers l'opérateur fautif. Enfin, la question du champ d'application de cette directive, aujourd'hui limitée aux comptes courants et dont la surtransposition pourrait amener à l'élargir aux comptes d'épargne et de crédit, est posée par les opérateurs de la qui souhaitent cet élargissement, alors que les banques sont partisanes du. Ainsi, la transposition de la directive dont il est question aujourd'hui, si elle est nécessaire, ne sera en tout état de cause pas suffisante pour encadrer l'évolution vertigineuse des nouvelles technologies appliquées à la finance.

Si nous sommes donc d'accord sur ce point, nous ne comprenons pas pour autant, nous non plus, que les agrégateurs de comptes, dont nombre d'entre eux proposent déjà aux consommateurs des offres de gestion de leur épargne ou de crédit, ne soient pas tenus de contracter une assurance de nature à rassurer le consommateur. Dans ce domaine, s'en remettre à une future directive européenne nous paraît en tout état de cause- cela a été dit par notre rapporteur général -extrêmement risqué. Si le Gouvernement considère, et on peut parfaitement l'admettre, que l'amendement voté à l'unanimité par la commission doit juridiquement être réécrit ou retravaillé,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, mes chers collègues, le présent projet de loi a pour objet de ratifier l'ordonnance portant transposition de la directive européenne concernant les services de paiement dans le marché intérieur. En ratifiant cette ordonnance, nous ferons oeuvre de modernisation de notre code monétaire et financier pour l'adapter aux évolutions de l'industrie financière et, surtout, à la numérisation de l'économie. Cette modification de notre droit est nécessaire à la fois pour l'activité des entreprises, mais également dans un souci de protection des consommateurs, de sécurité et de responsabilisation des acteurs financiers. Cette directive comporte trois dispositions essentielles, qui ont été rappelées. D'abord, elle pose les bases d'un droit d'accès aux comptes de paiement, en consacrant de nouveaux acteurs dans cette activité. Ensuite, elle renforce les normes de sécurité des données en rendant obligatoire l'authentification forte et en précisant les modes d'accès du client à son compte de paiement en ligne. elle consolide les droits des utilisateurs de services de paiement et améliore la supervision transfrontalière des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique. J'ajouterai que cette directive vise également à développer en France une pratique répandue en Europe, celle du, c'est-à-dire la possibilité de retirer des espèces chez un commerçant au moment d'un paiement. était théoriquement applicable en France mais, à défaut de cadre juridique prévoyant ses modalités d'application, il ne pouvait être mis en oeuvre. Le présent projet de loi, dans sa version issue de l'Assemblée nationale, prévoit ainsi d'autoriser mais aussi d'encadrer cette pratique du, notamment en fixant un montant maximal. C'est une bonne mesure, mais nous espérons que ce montant sera suffisamment élevé pour préserver l'intérêt du service pour le client, tout en permettant la prévention des risques. Tous ces éléments techniques sont importants. Ils permettent d'avancer vers un système financier européen et français plus performant et plus sûr. Je voudrais néanmoins évoquer à présent l'enjeu politique de ce texte et, en creux, ce qu'il révèle de la construction européenne. Nous avançons à grands pas vers l'Union des capitaux. La libre circulation des capitaux et des services financiers est une réalité, perfectible certes, mais c'est une réalité ! Sous la double influence des traités et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, toute mesure nationale dissuadant les mouvements de capitaux entre les États membres est désormais interdite. Mais qu'en est-il des citoyens européens ? L'Union des travailleurs, l'Union des étudiants, l'Union des artistes, l'Union des chercheurs sont-elles aussi complètes que l'Union des capitaux ? Les combats menés par la France et par une député européenne française courageuse, Élisabeth Morin-Chartier, sur la question des travailleurs détachés illustre la peine que nous avons à bâtir l'Europe sociale, c'est-à-dire, mes chers collègues, l'Europe des êtres humains. Je salue ainsi l'accord qui a été trouvé cette semaine sur la directive « travailleurs détachés » au Parlement européen. Nous nous rapprochons du principe élémentaire de justice « à travail égal, salaire égal, sur un même lieu de travail Je salue aussi la proposition de la Commission européenne de créer une « Agence européenne du travail » chargée de mieux contrôler la circulation des travailleurs, pour éviter le dumping social entre les États. Je salue enfin de manière générale, et mon groupe Les Indépendants avec moi, les mesures qui équilibrent l'intégration économique par une intégration sociale et culturelle. L'une ne va pas sans les autres, sous peine d'alimenter les accusations d'Europe à deux vitesses, Europe pour les élites, Europe pour les marchands. Je me permets cette digression- je m'en excuse, monsieur le rapporteur, mes chers collègues -sur ce projet de loi éminemment technique, afin de rappeler que, derrière la technique, il y a toujours de la politique, et que la politique consiste à faire des choix. Notre groupe Les Indépendants choisit un système financier plus sûr et plus moderne : nous voterons donc bien entendu en faveur de ce projet de loi. Mais nous choisissons également une construction

après le projet de loi relatif à la protection des données personnelles, dont nous avons débattu hier, nous examinons aujourd'hui un autre texte d'adaptation de notre droit aux évolutions technologiques liées au numérique, en l'occurrence dans le domaine financier. Notre Haute Assemblée est de plus en plus amenée à légiférer sur ces sujets. Le groupe du RDSE s'y intéresse et il est fier d'apporter, comme dans les autres domaines, sa pierre à l'édifice.

du coffre-fort numérique, que nous mettons désormais en pratique, mes chers collègues, avec l'application JULIA, de la déclaration des revenus des utilisateurs de plateformes, de la réglementation des jeux en ligne ou encore du passionnant débat d'octobre dernier sur l'intelligence artificielle. Après les excellentes interventions de mes collègues, que dire de plus, dans le temps imparti, sur la transposition de cette directive dite « DSP 2 », dont le niveau de technicité nous oblige, peut-être plus encore que d'habitude, à nous en remettre à l'expertise des rapporteurs ? Je m'intéresserai, dans un premier temps, à la procédure de transposition en tant que telle, puis, dans un second temps, au contenu de l'ordonnance et du projet de loi.

la précédente directive, dite « DSP 1 », avait déjà été complètement transposée, si bien que le travail de transposition était cette fois-ci plus limité. De fait, l'ordonnance ne comporte « que » 35 articles, alors que la directive dite « DSP 2 » en compte 117. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 13 janvier dernier, c'est-à-dire la veille de l'expiration du délai fixé. Ce caractère tardif de la transposition est peut-être dû au calendrier électoral particulièrement chargé de l'année dernière. Quoi qu'il en soit, on constate que la moitié environ des États membres, et non des moindres, n'ont pas encore pris de mesure de transposition. J'en viens maintenant au contenu du projet de loi. L'article 1 prévoit la ratification de l'ordonnance en tant que telle. Les articles 2 à 6 portent des rectifications, essentiellement techniques, à l'ordonnance. On ne peut que souscrire, dans les grandes lignes, aux mesures proposées

Je salue tout particulièrement l'abaissement de 150 à 50 euros de la franchise payée par l'utilisateur en cas de paiement non autorisé à la suite du vol, de la perte ou du détournement d'un instrument de paiement. Il s'agit d'une mesure de bon sens en faveur de la protection des consommateurs. L'article 1, ajouté à l'Assemblée nationale, encadre le, dont, je l'avoue, j'ai découvert l'existence et, surtout, l'évolution. Cette pratique, encore peu répandue en France il est vrai, pourrait se révéler utile, à condition d'être correctement encadrée, pour éviter les abus,

Je suivrai avec intérêt la publication du décret fixant notamment le montant maximal de retrait. L'article 1, également issu de l'Assemblée nationale, mais plus technique, concerne les mesures transitoires de communication entre prestataires de services de paiement et gestionnaires de compte.

en cas d'opération non autorisée, d'accès non autorisé ou frauduleux à ces données ou d'utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données. Bien qu'elle sorte du champ de la directive, cette mesure vise également à protéger les consommateurs face à des technologies qui se développent très rapidement. Elle nous paraît tout à fait judicieuse et pertinente.

en 4G ou en 5G et en très haut débit. Or, comme l'a fait remarquer mardi dernier, lors des questions d'actualité au Gouvernement, notre collègue le président Patrick Chaize, sur ce point, le Gouvernement semble avoir beaucoup reculé, notamment pour les populations les plus isolées.

Et je rappelle que, dans la querelle des anciens et des modernes, ce sont les anciens qui,, ont gagné ... L'essor des nouvelles technologies a favorisé l'émergence de nouveaux acteurs, tant pour l'initiation de paiement que pour l'information sur les comptes. Ces nouveaux acteurs permettent aux utilisateurs d'accéder aux données de l'ensemble de leurs comptes et produits bancaires et, surtout, d'initier des ordres de paiement, y compris sur les moyens d'épargne. Cela permet aussi aux, comme l'ont dit très bien précédemment un certain nombre de

Le nombre d'utilisateurs de ces nouveaux services a connu une croissance rapide, voire exponentielle- c'est la norme en matière de nouvelles technologies ! Comme l'a rappelé notre rapporteur, 4 millions de consommateurs ont déjà eu recours à un agrégateur de comptes et 2,5 millions ont déjà fait appel à un initiateur de paiement. Ce n'est pas rien ! Ce n'est plus un sujet médiocre aujourd'hui. C'est de nos, de notre système bancaire, mais avant tout de l'argent des Français qu'il s'agit. Ainsi, la directive permet de mettre en place des mesures de proportionnalité pour les acteurs réalisant de petits volumes de transaction et, en ce sens, de diminuer, de 150 à 50 euros, les seuils de franchise qui s'appliquent aux consommateurs subissant un préjudice.

de qui, dans un autre pays, agiraient dans des conditions peu conformes à l'intérêt des consommateurs. C'est le minimum ! La directive que nous transposons élève, en outre, les standards de sécurité pour les transactions. Une obligation d'authentification forte pour les paiements en ligne est ainsi prévue,

Les agrégateurs de comptes et initiateurs de paiement ont l'obligation de communiquer avec le gestionnaire de compte par le biais d'un canal de communication sécurisé et standardisé, afin de préserver la confidentialité des données bancaires et d'obtenir un agrément de Afin de faire face à d'éventuelles fraudes, une assurance doit être également souscrite par le prestataire, permettant de rembourser la banque si la responsabilité du prestataire est engagée. Un article a été introduit par nos collègues de l'Assemblée nationale, sur l'initiative du Gouvernement,

Ce service reposera, en outre, sur la base du volontariat et ne pourra évidemment pas être imposé à un commerçant. Enfin, l'Assemblée nationale a adopté, toujours sur proposition du Gouvernement- je tiens à le souligner un amendement tendant à ce qu'un décret définisse des modalités transitoires de communication entre les prestataires de services de paiement et les gestionnaires de compte, dans l'attente de l'entrée en vigueur, en septembre 2019, des normes techniques de de réglementation définissant les modalités de communication standardisée au niveau européen. On voit donc que le Gouvernement incite les assemblées à prendre des mesures transitoires, lorsque l'Union européenne les a oubliées. Tel était le sens de l'amendement de M. le rapporteur, adopté à l'unanimité des membres de la commission des finances : protéger le consommateur, dans l'attente

La Commission européenne a pris beaucoup de retard dans l'élaboration de la norme technique réglementaire devant préciser le fonctionnement de ces API. La directive prévoit une entrée en vigueur de ces dernières à l'été 2019 C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a souhaité que les dispositifs relatifs à la sécurité entrent en vigueur le plus tôt possible, afin de sécuriser ces données. D'ailleurs, tel est exactement le sens de l'amendement de M. le rapporteur général. Dans l'attente d'une solution européenne, la commission des finances a souhaité garantir la possibilité, pour l'utilisateur, d'obtenir un remboursement auprès du prestataire tiers en cas de fraude, la mise en place d'une obligation d'assurance complémentaire pour les comptes non couverts par la directive. La directive ne concerne, en effet, que les comptes de paiement. Or les nouveaux acteurs reconnus par la directive permettent aujourd'hui aux utilisateurs de passer des ordres et d'agréger les données concernant l'ensemble de leurs comptes et produits d'épargne. Les sommes en jeu sont considérables, car les personnes qui possèdent plusieurs comptes en banque

Dans ce contexte, pour la commission, s'il n'apparaît pas souhaitable d'étendre les dispositions de la directive à l'ensemble des comptes et produits d'épargne, ce chantier devant être mené au niveau européen, la question de la responsabilité en cas de fraude ne peut être laissée longtemps sans réponse.

Pour le reste, le texte ne pose pas de difficultés. Le groupe Les Républicains votera ce projet de loi de ratification, tel qu'il a été modifié par notre commission. La parole est à M. François Patriat, pour le groupe La République En Marche.

le projet de loi de ratification d'une ordonnance d'apparence technique, laquelle transpose la directive dite « DSP 2 », relative aux services de paiement dans le marché intérieur. Ce texte est nécessaire, en premier lieu, parce qu'il régule une activité encore mal encadrée et qui correspond à une demande sociale. Le premier apport de la directive est, en effet, de reconnaître de nouveaux acteurs qui interviennent entre les banques et leurs clients, qui rendent de nouveaux services et qui facilitent les paiements. Il s'agit des agrégateurs de comptes, utiles pour les particuliers que nous sommes comme pour les entreprises, auxquels ils offrent un accès pédagogique à leurs informations financières. Le client de ces services a ainsi une vision consolidée de ses comptes sur une seule interface. Il s'agit aussi des initiateurs de paiement, dont l'activité d'intermédiaire doit permettre de fluidifier la réalisation des virements. Ce service est très développé en Allemagne, où le paiement en ligne par carte est moins naturel. En reconnaissant ces activités, madame la secrétaire d'État, la directive renforce les garanties pour les usagers elle impose une couverture par une assurance de responsabilité civile professionnelle, mais elle durcit aussi les conditions d'agrément et de supervision des établissements de paiement. Les pouvoirs des superviseurs, comme l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en France, sont élargis. La directive renforce également la supervision transfrontalière des établissements de paiement : elle prévoit un mécanisme d'échange d'informations entre les autorités de supervision et accroît les échanges dans le cadre de la surveillance des établissements de paiement. Elle permet ainsi de lutter contre le risque de. Enfin,

la directive accompagne une évolution sociale et technologique, réglemente un secteur qui se développe et harmonise la réglementation. Nous pouvons nous enorgueillir que la France fasse le choix d'une transposition rapide

Dans une économie de services où l'activité est facilement délocalisable, l'amendement de la commission des finances sur l'utilisation fraudeuse des données non couvertes par la directive montre le besoin d'une couverture uniforme par des règles européennes. Je salue Je salue la disposition, ajoutée dans le projet de loi par un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, qui prévoit l'accompagnement du. Ce service, qui existe, par exemple, au Canada, en Allemagne ou au Royaume-Uni, permet aux commerçants de rendre du liquide aux clients qui ont payé par carte. Pour les commerçants, le présente un double avantage : c'est un nouveau service à offrir, ainsi qu'un moyen de gérer plus efficacement leurs encours en caisse. C'est aussi un avantage pour les consommateurs, notamment pour accéder aux espèces dans les lieux trop éloignés des guichets. On sait que le mouvement de suppression des guichets physiques par les banques dans nos territoires est réel

Mon avis est que cette directive est politique. Elle est politique, parce qu'elle complète l'édifice qu'est le marché intérieur. Elle est politique, parce qu'elle donne des garanties aux citoyens européens. Elle est politique, parce qu'elle harmonise des réglementations dans un secteur en plein essor. Soyons réalistes beaucoup des critiques adressées à l'Union européenne, sur la concurrence fiscale par exemple, viennent d'un manque d'harmonisation des réglementations au niveau européen qui est le fait non de l'Union européenne en tant qu'entité abstraite, mais des États membres.

2. Cet amendement vise à protéger le consommateur. Nous rejoignons bien évidemment la préoccupation de la commission des finances,

la perplexité et les nombreuses questions qu'a soulevées l'examen de cette proposition de nouvel article.

protection proposée nous a gênés : certains agrégateurs ne seraient pas couverts, en particulier ceux qui décideraient de ne pas accéder aux comptes de paiement et donc de ne pas demander d'agrément. Ils pourraient alors proposer une agrégation sur tous les autres comptes, sans obligation d'assurance. De même, les acteurs qui choisiraient de se faire agréer dans un autre État membre que la France

Nous souhaitons engager une mission de réflexion permettant d'associer les acteurs de façon très précise et technique afin de formuler des propositions à porter auprès de la Commission européenne. Cette mission toute mesure transitoire pertinente à adopter au niveau national. J'insiste sur la complexité du sujet, sur la nécessité d'analyser les impacts industriels que pourraient engendrer l'intervention de ces nouveaux acteurs et le développement de nouveaux modèles économiques dans les segments de l'épargne et sur le fait que cet effort de sécurisation

Je comprends que vous considériez que le temps de la négociation européenne n'est pas compatible avec celui, plus rapide, de l'avancée des usages qu'offre la technologie. À défaut de partager votre enthousiasme pour la solution technique suggérée, je rejoins votre souci de sécurisation des consommateurs. Aussi, à ce stade de la procédure parlementaire, le Gouvernement retire son amendement de suppression. Très bien

Ces dispositions trouvent en particulier à s'appliquer dans le cas des comptes de cantonnement ouverts par ces établissements sur lesquels ils déposent les fonds reçus de leur propre clientèle. Une incertitude existe en effet sur le fait que la délégation conférée au ministre chargé de l'économie au a) du 10° de l'article L. 312-16 de préciser par voie d'arrêté « les conditions dans lesquelles l'ayant droit de tout ou partie des sommes figurant sur un compte, qui n'est pas le titulaire nominal, peut bénéficier de la garantie des dépôts » couvre ce cas de figure, la loi ne prévoyant de dérogation expresse qu'en ce qui concerne les comptes ouverts par les entreprises d'investissement.

cas de défaillance d'un établissement de crédit, ces comptes puissent bénéficier de la garantie des dépôts au même titre que les clients des entreprises d'investissement dont les fonds sont également déposés sur un compte de cantonnement. Dans l'hypothèse inverse, la défaillance d'un établissement de crédit teneur de compte entraînerait des effets de contagion sur les établissements de paiement, entraînant probablement leur propre défaillance et leur incapacité à restituer à leur clientèle- généralement constituée de particuliers -les fonds qu'ils ont collectés. Cela conduirait à rendre inefficaces les mesures de protection, en particulier de cantonnement des fonds, dont ils sont censés bénéficier au regard des textes applicables, notamment européens. Quel est l'avis de la commission ? Après les propos tenus sur l'amendement précédent, vous vous en doutez, la commission est évidemment très favorable à cet amendement, qui va dans le sens de la protection du consommateur. Il s'agit davantage d'une clarification que d'une véritable innovation.